l'enseignement professionnel est une voie importante de notre système éducatif. Pourtant, cette filière a perdu 100 000 élèves en vingt ans et ses résultats pour l'obtention d'un emploi sont décevants. deux ans après avoir obtenu leur diplôme, seuls 41 % des titulaires d'un CAP et 51 % des bacheliers professionnels ont trouvé un emploi. Pour nombre de jeunes, l'enseignement professionnel est vécu comme une voie de relégation, une sanction pour leurs difficultés scolaires, une filière de l'échec.

vers un lycée professionnel et plus de la moitié des lycéens de cette filière viennent de quartiers défavorisés, selon une étude réalisée par Sciences Po. Un tiers des élèves de l'enseignement professionnel sont boursiers, fois plus élevée que dans l'enseignement général et les enfants de cadres ne représentent que 7 % des effectifs de la voie professionnelle. L'éducation nationale a une responsabilité en la matière,

Il est également incontestable que trop de jeunes suivent des formations qui ne débouchent pas sur un emploi après le bac. Ainsi, 60 % des « lycéens professionnels » sont scolarisés dans les filières tertiaires du bac professionnel, alors que ces filières recrutent au niveau bac+2. Plus largement, les effectifs sont surtout concentrés en commerce et vente et en sanitaire et social, alors que, mis à part l'aide à domicile et l'hôtellerie et la restauration, les pénuries de compétences se focalisent aujourd'hui dans l'industrie.

Ainsi, au lycée Éric-Tabarly des Sables-d'Olonne, où s'exprimait, le 13 septembre dernier, le Président de la République, on trouve en effet des formations « insérantes », telles que la chaudronnerie ou la maintenance nautique, preuve que le système abrite aussi de réelles pépites.

La réforme de 2019 n'entendait-elle pas déjà favoriser les synergies entre la voie scolaire et le monde de l'apprentissage, afin que les deux systèmes jouent la carte de la complémentarité ? selon les termes mêmes du ministre d'alors, de transformer les établissements professionnels en « Harvard professionnels » ? Cette ambition semble avoir tourné court Pourtant, alors même que la réforme de 2019 n'a pas été analysée, les annonces faites par le Président de la République fixent déjà un cadre précis : doublement des heures de stages, révision de la carte des formations, réorientation des enseignants et recrutement d'un personnel issu du monde professionnel. Après avoir annoncé ces mesures très précises, le président Emmanuel Macron a maintenant recours à une série de débats calqués sur le modèle du Conseil national de la refondation ; on peut s'interroger sur la méthode

Comment mieux préparer la poursuite des études dans le supérieur ? Comment améliorer le taux d'accès à l'emploi ? Et comment donner des marges de manoeuvre aux établissements, tout en conservant le caractère national des diplômes ? Ces groupes, composés de représentants des syndicats, des régions, des parents d'élèves, des établissements, des entreprises ou encore des collectivités, sont pilotés par un recteur accompagné d'un inspecteur général. Après les inquiétudes provoquées par les réformes annoncées par le chef de l'État aux Sables-d'Olonne, on comprend que le Gouvernement tâche, manifestement, de rassurer. Toutefois, les principaux syndicats d'enseignants, qui dénoncent un passage en force, ont refusé de participer à ces groupes de travail. Une mobilisation a eu lieu le 18 octobre dernier et elle doit être renouvelée cette semaine. Elle traduit les difficultés de mise en oeuvre des pistes proposées par le chef de l'État. La double tutelle exercée dorénavant sur la réforme des lycées professionnels par les ministères chargés du travail et de l'éducation nationale est également l'objet d'inquiétudes. Certains y voient le renforcement bénéfique du lien entre le lycée professionnel et le marché du travail

trancher ce débat, en observant simplement les évolutions des différents pays, on constate que les formations professionnelles de qualité reposent sur un solide socle commun de culture et de compétence générales. il s'agit d'une condition pour accéder aux études supérieures après le bac pro. Quel que soit le point de vue et sans anticiper le débat que nous aurons tout à l'heure, le sujet sensible de la durée des stages soulève de nombreuses questions. C'est à travers celles-ci que l'on peut aborder le sujet sans préjugé ni tabou : comment trouver assez d'entreprises pour accueillir les élèves, alors que c'est déjà une difficulté ? Faut-il proposer des incitations aux entreprises pour ouvrir un vivier d'offres ? Les lycéens percevront-ils une rémunération versée par l'État, comme cela a déjà été évoqué ? Le rapprochement avec le monde professionnel impliquera-t-il pour les lycées de recruter davantage de professeurs associés issus des entreprises ? Ce rapprochement passera-t-il par une participation accrue à la gouvernance des conseils d'administration des lycées ? N'est-il pas indispensable de mieux adapter la carte des formations aux réalités économiques, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des diplômés ? Dans ce cas, comment organiser la reconversion des enseignants ? Enfin- au Sénat, je serais tenté de dire « d'abord » -, comment mieux associer les collectivités, qui sont les mieux à même de faire le lien entre les besoins des entreprises et l'offre de formation On le voit, les questions sont nombreuses, mais tous les efforts seront vains si nous ne parvenons pas à établir l'image d'un enseignement professionnel adapté tant aux élèves et à leurs difficultés qu'aux besoins de secteurs économiques d'avenir. Le groupe Les Républicains souhaite que le présent débat contribue à éclairer la voie à suivre, tant par ses questionnements que par ses propositions, et que le Parlement soit associé à cette rénovation indispensable.

je salue le choix du groupe Les Républicains d'avoir proposé ce débat consacré à l'enseignement professionnel. Nous pensons tous, au sein de cet hémicycle, qu'il est nécessaire de faire reconnaître l'enseignement scolaire professionnel comme une véritable voie de réussite aux yeux des jeunes,

de 800 000. Cela correspond à deux ou trois fois le nombre d'apprentis que comptait notre pays en 2018. L'essor considérable de l'apprentissage a contribué à faire diminuer le taux de chômage des jeunes de manière durable, en le situant à 15,9 %.

La situation actuelle est source de frustrations tant pour les jeunes et leurs familles que pour les enseignants eux-mêmes. L'impression d'être déclassé, méprisé par un système qui semble punir les enfants en difficulté nourrit le ressentiment et l'échec. ressentiment et l'échec. Des transformations de la voie professionnelle ont déjà été accomplies lors du précédent quinquennat, dans le contexte pourtant difficile de la crise sanitaire. Cette première transformation fournit un socle sur lequel nous devons continuer de bâtir pour aller plus loin, dans le cadre d'un investissement structurel et résolument tourné vers la réussite des élèves. C'est notre responsabilité à tous : rétablir l'ascenseur social pour ces jeunes et permettre de rendre tangible l'égalité des chances pour les publics les plus fragiles. Les lycées professionnels, on le sait trop peu, accueillent un tiers des jeunes lycéens en France, qui sont souvent des enfants cumulant des vulnérabilités scolaires et sociales. les 627 000 « lycéens professionnels » sont majoritairement issus de milieux défavorisés et se retrouvent souvent en situation d'échec pendant ou après leur scolarité. Voici quelques données pour vous en convaincre : 33 % de ces élèves sont issus d'une famille ouvrière et 3 % d'une famille de cadre une forte proportion est issue de l'immigration ou est allophone ; 5 % des élèves sont en situation de handicap, contre 1 % des « lycéens généraux

En outre, l'organisation pédagogique actuelle ne prend pas suffisamment en compte les mutations économiques, les réalités des difficultés des élèves et les défis du territoire. Elle ne s'adapte pas non plus suffisamment aux trajectoires et aux profils des élèves.

la carte des formations est parfois déconnectée des enjeux du marché du travail : de nombreuses formations tertiaires ne sont pas suffisamment « insérantes » ; les investissements dans les plateaux techniques et les efforts déployés pour la reconversion des enseignants se révèlent souvent mal connectés aux réalités économiques. la préparation au monde professionnel n'est pas satisfaisante et n'offre pas aux jeunes la maîtrise nécessaire des codes de l'entreprise ou des techniques de recherche d'emploi pour s'insérer efficacement dans le monde du travail.

l'offre de formation préparatoire aux études supérieures, du type « mention complémentaire » ou « diplôme de spécialité professionnelle » en une année, est insuffisante. Dans ce contexte, nous nous sommes assigné trois objectifs clairs pour réussir cette réforme, que nous allons bâtir avec l'ensemble des acteurs concernés. concernés. Premièrement, nous souhaitons réduire le nombre de décrocheurs, éviter cette fuite des élèves qui ne trouvent pas leur place en lycée professionnel. Entendons-nous bien personne n'accuse les lycées professionnels d'être la cause unique du décrochage ; ils en sont souvent le réceptacle, héritant de difficultés liées à la fois aux fragilités personnelles des élèves et au manque de souplesse des parcours de formation.

investir dans les lycées professionnels comme jamais auparavant. C'est la première fois qu'un Président de la République apporte un tel soutien, lors d'une campagne et dans son projet présidentiel,

qui soient plus en phase avec la préparation des grands défis collectifs de demain. Je pense évidemment aux transitions écologiques et numériques, mais également à la révolution de la longévité, c'est-à-dire aux enjeux du vieillissement de la population, au défi de la transition vers une société plus inclusive et plus et plus solidaire, qui passe par un meilleur accompagnement du handicap dans tous les secteurs, ainsi qu'à notre politique de souveraineté économique et de réindustrialisation du pays. La multiplication des périodes de formation en milieu professionnel- les stages -, combinée à la gratification des élèves pendant ces périodes, doit permettre de rapprocher encore davantage le lycée professionnel du monde de l'entreprise et de conforter la motivation des élèves ainsi que leur engagement à réussir. Les stages contribuent à donner du sens, de l'expérience et des contacts, ils renforcent

est à M. Pierre-Jean Verzelen. Madame la ministre, vous l'avez indiqué, l'apprentissage connaît un succès sans précédent. En période de crise pandémique, le nombre d'apprentis a été multiplié par deux, pour atteindre aujourd'hui 740 000. Même si ces chiffres doivent se confirmer dans le temps,

ensuite, lorsque l'on fait preuve de volonté politique et que l'on met les moyens en face, les résultats sont là ; enfin, quand c'est attractif pour l'entreprise et pour le jeune, notamment en matière d'embauche et de débouchés, cela fonctionne. La question qui se pose maintenant est : comment l'enseignement professionnel peut-il connaître le même élan ? Certes, les problématiques sont différentes, mais nous devons pouvoir créer des synergies entre ces deux voies. L'une des leçons de l'apprentissage est que les formations se sont adaptées aux bassins d'emploi et aux réalités des territoires, et pour cause : les jeunes, les entreprises et les centres de formation disposent de marges de manoeuvre pour s'organiser. Nous avons donc besoin, là encore, de liberté et de souplesse. L'une des difficultés de l'enseignement professionnel réside dans le manque de débouchés concrets moins d'un élève sur deux a trouvé un emploi douze mois après sa sortie de formation, alors que ce taux atteint quasiment 70 % chez les apprentis.

Allez-vous accorder plus d'autonomie aux chefs d'établissement, afin de leur permettre de s'adapter au mieux aux besoins et aux réalités de leur bassin d'emploi ? La parole est à Mme la ministre

le Président de la République a évoqué, le 13 septembre dernier, les grands axes de la réforme des lycées professionnels : rapprocher les lycées professionnels des entreprises, fermer certaines formations et en ouvrir d'autres, le tout en lien avec les régions, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Autant de bon sens serait louable s'il ne se bornait pas à décrire l'existant ... En effet, le lycée des métiers de la mer et de l'espace de Gujan-Mestras, près d'Arcachon, ne traite pas de la montagne et les lycées des métiers du bois se trouvent déjà dans des régions forestières, comme les Landes. Ce qui relève moins du bon sens en revanche, c'est la tendance au détricotage de l'enseignement professionnel dans le secondaire, dans laquelle s'inscrit cette réforme : moins d'établissements, moins d'élèves, moins d'heures d'enseignement, moins de moyens, moins d'enseignants. Hélas, cette logique n'a pas disparu des objectifs des groupes de travail mis en place à la suite de la mobilisation exceptionnelle, le 18 octobre dernier, des professeurs de lycée professionnel et des syndicats. Aujourd'hui, plus de 26 % des lycéens obtiennent un bac professionnel et, pourtant, ils ne représentent que 6 % des étudiants à l'université et 17 % des À côté de leur connaissance plus précoce du monde de l'entreprise, les lycéens de ces filières doivent pouvoir bénéficier d'un socle d'enseignement général leur permettant de prétendre, si telle est leur ambition, à des cursus dans le supérieur. C'est le cas de la moitié d'entre eux aujourd'hui ; je pense notamment aux écoles supérieures de journalisme et de communication, qui accueillent dans leurs murs des titulaires d'un bac pro en artisanat et métiers d'art avec une option communication visuelle plurimédia, tant l'agilité numérique et technique est devenue capitale pour ces filières. pensez-vous sincèrement que la réforme que vous entendez mettre en place donne aux bacheliers professionnels une chance égale d'accéder à des formations supérieures en adéquation avec leurs aspirations personnelles ?

à 2020. Néanmoins, un problème demeure : ces jeunes se heurtent souvent à des difficultés pour trouver leur stage, leur alternance ou leur apprentissage dans une entreprise qui leur fera confiance.

Juste après l'obtention du CAP ou du bac pro, ces sorties rapides ne sont pas toujours couronnées de succès, puisque seulement 32 % de titulaires du CAP et 45 % des titulaires du bac pro trouvent un emploi dans les douze mois qui suivent Madame la ministre, il y a, à l'évidence, des marges de progrès pour améliorer la recherche d'emploi de ces jeunes, qui souhaitent entrer rapidement dans la vie active. Quelles pistes envisagez-vous pour leur permettre de trouver plus facilement un emploi et quels leviers pourraient inciter les entreprises à les recruter

ma part, sur la volonté du Président de la République d'adapter l'offre de formation des lycées professionnels aux besoins des bassins d'emplois locaux. S'il s'engage dans cette voie, le lycée professionnel verrouillera le destin des élèves qui en fréquentent les bancs, puisque leur appartenance géographique à cet instant déterminera leur carrière professionnelle. Alors qu'il faudrait, au contraire, veiller à ne fermer aucune porte à ces élèves, y compris dans l'accès à des études supérieures, on réduit leur capacité de choisir librement leur avenir, d'autant que la réforme prévoit également la diminution des heures consacrées aux enseignements fondamentaux. cette vision de court terme ne prend pas en compte la diversité des territoires. Qu'en sera-t-il de ceux où les bassins économiques sont fortement sinistrés et l'accès à l'emploi déjà compliqué ? En outre, cette vision fait peser sur les établissements et les professeurs dont la formation ne serait plus jugée adaptée la lourde charge de la reconversion pour répondre à ces nouveaux besoins, peut-être éphémères. Enfin, elle interroge sur la philosophie même de notre école. Le seul rôle de notre lycée professionnel serait-il de fournir une main-d'oeuvre prête à l'emploi pour les entreprises locales ? Pour conclure, les alertes que je vous lance sont partagées par les parents d'élèves et par les syndicats, attachés, comme nous devrions toutes et tous l'être, à la dimension nationale du bac professionnel et à la garantie de l'égalité entre les élèves. En tiendrez-vous compte dans le cadre des groupes de travail que vous avez réunis pour élaborer cette réforme ?

alors même que les élèves de l'enseignement professionnel ont besoin des enseignements généraux, car ils en sont souvent les plus éloignés ? Comment ceux qui le souhaitent pourraient-ils poursuivre des études supérieures à l'issue d'un tel cursus ? Et comment envisager envisager sérieusement une augmentation significative des périodes en entreprise quand on sait la difficulté de trouver des terrains de stage ? Vous dites vouloir augmenter la rémunération des stages pour l'aligner sur celles des apprentis.

Les élèves des lycées professionnels, qui représentent un tiers des lycéens de notre pays, méritent d'être traités à égale dignité de ceux de la voie générale. Enfin, depuis juin dernier, un décret permet aux enseignants des lycées professionnels d'enseigner en lycée général et technologique ou en collège, avec l'avantage que ceux-ci dispensent deux matières différentes. Cette réforme serait-elle une manière inavouée de faire face à la crise de recrutement que nous connaissons dans l'éducation nationale en raison de la faiblesse des salaires

et « mieux » sur les formations professionnelles. Les établissements vendéens avec lesquels j'ai pu échanger partagent le même constat : faute d'information, les débouchés multiples des lycées professionnels ne sont absolument pas valorisés, alors même que les choix en matière d'études supérieures et de passerelles ne manquent pas, allant du certificat de spécialisation à l'école d'ingénieur, en passant par le BTS, le bachelor Comment prôner et encourager l'excellence des filières professionnelles si nos jeunes n'ont pas de visibilité sur le « post-bac pro » et qu'ils n'ont pas conscience de la possibilité de poursuivre des études au-delà du lycée ? Madame la ministre, qu'entendez-vous faire pour offrir aux élèves et aux familles, mais également aux professeurs et aux établissements du secondaire, l'accès à une information complète et qualitative pour une orientation éclairée ? Orientation rimant avec affectation, j'aborderai également ce sujet. Actuellement, le service en ligne Affectation, accessible aux élèves de troisième, repose uniquement sur un arbitrage basé sur les résultats académiques obtenus par les élèves au cours de leur scolarité, sur la décision d'orientation prise au conseil de classe de fin de troisième et sur le nombre de places disponibles. L'intérêt et l'appétence des élèves pour la filière à laquelle ils candidatent ne sont pas pris en compte. Aussi, madame la ministre, que comptez-vous mettre en place pour intégrer le projet professionnel de chaque élève au système d'affectation ? La parole

que j'ai déjà cités. Un troisième enjeu touche précisément à la carte des formations. Un travail sur le choix de chacune des formations proposées et sur l'employabilité à l'issue de l'obtention du diplôme doit être mené, en collaboration

sous-valorisé, à tort. Pourtant, je rappellerai que, en marge de la voie professionnelle classique, le fameux compagnonnage français est inscrit depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité sous le titre « Le compagnonnage, réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier ». Pour peu qu'ils soient bien mieux reconnus socialement, comme ce fut le cas durant la pandémie avec les professions dites de première ligne, tous les métiers ont du sens. L'enseignement professionnel offre un potentiel de parcours nécessaires pour répondre à la fois aux aspirations de nombreux jeunes et aux besoins non satisfaits du marché du travail. Dans ces conditions, la réforme du lycée professionnel met davantage l'entreprise au coeur de la formation, notamment du projet de développement de l'apprentissage dans tous les secteurs d'activité et tous les lycées professionnels. Néanmoins, je m'interroge sur la tendance à une forte spécialisation de la voie professionnelle. En effet, il est observé que deux tiers se concentrent dans trois spécialités du secteur tertiaire : le commerce, la gestion-administration et les soins et services à la personne. En outre, le monde économique exprime, en son sein, une demande contradictoire. Certaines entreprises souhaitent des profils aux compétences transversales tandis que d'autres souhaitent que davantage de spécialités soient proposées aux élèves. Aussi, madame la ministre, comment résoudre cette équation entre de nouveaux besoins de spécialités, notamment sous l'effet des évolutions technologiques et industrielles, et une orientation des élèves vers un même type de formation ? La parole est à Mme la ministre

Madame la ministre, je vais vous donner l'occasion de répondre aux demandes de précisions de Mme Brulin. Ah ! En effet, je souhaiterais que vous reveniez sur la place des enseignements généraux dans la formation des jeunes en lycée professionnel. Concrètement, que fait-on ? peut se comprendre pour rapprocher formation en lycée professionnel et monde de l'entreprise, comment y parvenir sans réduire à la portion congrue la maîtrise des savoirs fondamentaux pour des élèves qui ne les maîtrisent qu'imparfaitement ? Tout à fait ! L'enjeu, pour ces élèves, est celui de la réussite professionnelle.

? En outre, réfléchissez-vous à la nature de ces enseignements généraux ? Ne faut-il pas renouveler leur contenu et leur didactique afin que les élèves ne les vivent pas comme la suite de leur scolarité marquée par l'échec, comme un nouveau point de départ ? Face à un tel objectif, ne faut-il pas étudier ce que font les lycées agricoles, lesquels organisent avec succès un enseignement socioculturel mêlant éducation à l'environnement social et culturel, éducation artistique, formation à l'autonomie et à la communication ? Madame la ministre, le renouvellement des enseignements généraux et des pratiques est-il à l'ordre du jour de vos concertations ? L'expérience des lycées agricoles peut-elle être élargie ? En somme, quelle est votre réflexion sur la place de l'enseignement des disciplines non professionnelles ? Très bien ! La parole est à Mme la ministre

De fait, les CAP et les bacs pro sont des diplômes professionnels à insertion professionnelle directe pour ceux qui le souhaitent, même si- nous l'avons dit -le taux d'accès à l'emploi après le diplôme doit être amélioré. Plus un jeune Plus un jeune fréquente l'entreprise, plus il a de chances de s'y insérer durablement. Nous devons le prendre en considération. Pour les élèves en CAP, l'enseignement professionnel représente 55 % du

cours des trois années de formation. J'aimerais vous rassurer. Nous préserverons le temps des savoirs fondamentaux : la réforme que nous menons n'a pas pour objectif de réduire le volume d'enseignement en lycée professionnel, qu'il soit général ou à caractère professionnel. S'il faut davantage de temps à ces lycéens pour qu'ils s'immergent plus et mieux

... Je regrette que vous n'ayez pas non plus répondu sur le contenu de ces enseignements généraux, qui a besoin d'être rénové. Voilà un beau sujet pour vos groupes de concertation.

Il n'est plus tolérable que ces établissements qui accueillent près d'un tiers des lycéens et des lycéennes de notre pays soient perçus comme une voie de garage, ou la destination des élèves en échec scolaire. L'urgence est à la revalorisation de ces formations, afin qu'elles soient perçues comme des lieux de réussite, de découvertes, de passions ou d'innovation. Or, depuis les annonces du Président de la République, on ne nous parle que de courbes du chômage, de taux d'employabilité, de taux d'insertion, mais aussi d'un allongement- largement évoqué par mes collègues -de 50 % des périodes de stage que personne ne demande Vous faites comme si la formation elle-même, voire les enseignants, était en cause, et la convergence avec l'apprentissage la seule issue. Or, pour beaucoup, les élèves qui arrivent en filière professionnelle ont vécu une orientation subie. Ils arrivent brisés par le système scolaire. C'est au contact de leurs enseignants qu'ils reprennent confiance, avec des parcours exemplaires d'étudiants devenus expert immobilier, conseillère bancaire, d'autres ouvrant leur propre boutique ou poursuivant des études en art ou en audiovisuel. reprise de confiance : les horaires excessifs, le travail de nuit, l'exposition aux produits toxiques voire le harcèlement sont trop souvent le quotidien de stagiaires perçus comme une main-d'oeuvre gratuite.

les heures d'enseignements généraux, qui permettent à ces enfants de s'émanciper et de choisir leur destin. Je vous demande enfin d'ouvrir de nouvelles filières dans les métiers d'avenir, ceux du numérique, des médias ou du développement durable.

Cet exemple n'en est qu'un parmi tant d'autres, car le désarroi est grand dans les différentes filières. Aussi, madame la ministre, ma question est double. Quel bilan tirez-vous de la transformation de la voie professionnelle menée par Jean-Michel Blanquer en 2019 ? Blanquer en 2019 ? À l'heure où l'on parle de faciliter l'accès de certains immigrés à des métiers dits en tension, pourquoi n'a-t-on pas prévu des structures de formation professionnelle ? Nous

vie. Comparaison n'étant pas raison, sans vouloir faire de généralités, donnons le salaire d'un façadier en début de carrière : environ 2 000 euros mensuels net.

a été déployée dans tous les lycées professionnels, et ce malgré la crise sanitaire. J'en remercie chaleureusement l'ensemble des personnels éducatifs et enseignants, dont je connais l'investissement en la matière. Cette transformation innovations pédagogiques. Je pense notamment à la co-intervention, qui est bien installée et produit des résultats de qualité. Elle permet de renforcer le nombre d'heures à effectifs réduits et d'associer plus étroitement enseignements généraux et enseignements professionnels de spécialité.

Plus des trois quarts des lycéens en situation de handicap sont scolarisés dans la filière professionnelle, alors que les lycées professionnels ne représentent que 30 % des effectifs de l'ensemble des lycées. Une telle disproportion alimente bien évidemment l'idée d'une voie plus subie que choisie.

La raison affichée par les employeurs est bien souvent la crainte de ne pas pouvoir accueillir et encadrer convenablement ces travailleurs. L'entrée dans l'entreprise d'une personne en situation de handicap par le biais d'un stage est une réelle opportunité d'insertion. est toutefois difficile pour ces jeunes, encore plus que pour les autres lycéens professionnels, de trouver une structure pour les accueillir. Ainsi, madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer si le cas particulier des lycéens en situation de handicap sera pris en compte au sein des fameux fameux groupes de travail que vous avez constitués ? Dans un contexte où de nombreux lycéens rencontrent déjà des difficultés pour trouver un stage en lien direct avec le métier auquel ils se forment, prévoyez-vous des mesures spécifiques afin que les lycéens fragilisés par le handicap puissent trouver des entreprises pour les accueillir ? La parole est à Mme la ministre

par un groupe de travail. Les enseignants des lycées professionnels, comme l'ensemble des autres enseignants, sont formés à la pédagogie adaptée aux élèves en situation de handicap. Nous souhaitons poursuivre et accentuer la formation continue, car il

national de l'accès aux formations professionnelles pour les jeunes, mais aussi des diplômes professionnels. Je ne reviendrai pas non plus sur votre volonté d'hyperspécialiser les élèves des lycées professionnels, en lien avec les besoins immédiats des entreprises locales. Je rappelle que les élèves des lycées professionnels comme tout autre lycéen ou lycéenne, d'acquérir des savoirs fondamentaux. Or ces acquisitions ont déjà été fragilisées par la réforme Blanquer. Les élèves doivent pouvoir bénéficier d'heures d'enseignement, dans les disciplines tant générales que professionnelles, notamment pour améliorer leur réussite aux examens. Des jeunes qui entrent en CAP ou en bac pro à 14 ans ou 15 ans ont besoin d'être encadrés par les professionnels de l'éducation que sont leurs professeurs Avec un accroissement de 50 % du temps dédié aux stages professionnels, cette réforme entraînera inévitablement une diminution des heures d'enseignement et les suppressions de postes qui vont avec,

et ouvre le marché des formations aux filières et à un très grand nombre d'opérateurs. Le développement de l'apprentissage, qui a presque doublé en quatre ans, a été rendu possible par la libéralisation du système et par la mise en place de fortes incitations financières pour les entreprises accueillant un apprenti : prime exceptionnelle de 5 000 euros à 8 000 euros selon l'âge et exonération des charges. 2022, en Normandie, on dénombrait 120 centres de formation, contre 59 en 2018. Cependant, cette évolution, qui permet de répondre en partie au besoin des entreprises, a profondément transformé l'équilibre des formations sur notre territoire et posé la question de la concurrence entre établissements de formation professionnelle.

Contrairement à l'apprentissage, qui, longtemps dévalorisé, redevient une formation initiale reconnue, les lycées professionnels n'ont pas réussi à convaincre de l'excellence de leur enseignement et peinent à recruter. Ces établissements, déjà présents sur nos territoires, devraient pourtant être complémentaires avec d'autres centres de formation et non en concurrence directe. Alors, madame la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour en finir avec la concurrence entre CFA et lycées professionnels, et pour que, enfin, la filière de l'enseignement professionnel redevienne attractive ? La parole

pas les mêmes profils de jeunes, qui sont à des étapes différentes de leur vie et n'ont souvent pas le même niveau de diplôme. Le Gouvernement cherche à construire avec tous les acteurs concernés une réforme de l'enseignement professionnel visant à sécuriser les parcours des jeunes, en permettant

le renforcement des enseignements au lycée professionnel et l'intensification de l'accompagnement. À cet égard, il n'existe aucune concurrence entre apprentissage et lycées professionnels. D'ailleurs,

À moins de surcharger les semaines, cette augmentation du temps passé en stage impliquera une diminution des heures d'enseignement général et professionnel français, mathématiques, mais aussi gestion et économie, autant d'enseignements qui doivent être dispensés pour préparer ceux qui le souhaitent à un cursus dans l'enseignement supérieur.

et d'une culture générale, sans omettre l'indispensable apprentissage du français et des langues vivantes, constituent des préalables impératifs à la cohésion de notre société. L'équation est donc la suivante : comment augmenter les périodes de formation sans toucher aux volumes horaires des enseignements généraux et professionnels ? Si une certaine autonomie dans la vie de ces établissements peut être bénéfique, l'organisation locale des heures d'enseignement ne risque-t-elle pas de remettre en cause le caractère national du diplôme ? La réforme fait actuellement l'objet d'une concertation, lancée le 21 octobre dernier. Je ne veux donc pas préjuger des conclusions que vous en tirerez, mais je tiens à vous interpeller et à entendre votre avis sur ce sujet préoccupant, à savoir les conséquences de la diminution du temps scolaire sur l'avenir de nos lycéens.

soulève la question du pilotage de la réforme et de son financement puisque les ministères de l'éducation nationale et du travail sont appelés à collaborer, qui pourrait se révéler compliqué. La rémunération des élèves sera-t-elle assurée par les entreprises ? Une partie sera-t-elle prise en charge par l'État ? quel ministère sera concerné ? La question du choc de l'offre pour les stages est aussi un motif d'inquiétude. S'il a été démontré qu'il existe une synergie entre les lycées professionnels et les entreprises locales dans les villes moyennes, la situation est beaucoup plus inquiétante à l'échelle des grandes agglomérations. À cela s'ajoute l'éventuelle concurrence avec l'apprentissage, dans un tissu d'entreprises en nombre limité. Entendez-vous établir une cartographie des bassins d'emploi et y associer les élus ? Lors de la présentation de la réforme au mois de septembre, le Président de la République a expliqué que « cette réforme [entrerait] en vigueur de manière très progressive ». Toutefois, l'inquiétude ne faiblit pas. Une nouvelle journée de mobilisation nationale est d'ailleurs prévue cette semaine, le 17 novembre. Faute de fournir une feuille de route aux enseignants, pouvez-vous enfin leur apporter des réponses précises ?

lucides sur les constats et que nous sommes bien évidemment engagés dans une démarche d'investissement et de coopération avec les acteurs.

Dévalorisé, peu plébiscité par les parents dans l'Hexagone, l'enseignement professionnel est encore fortement associé à la faiblesse des résultats scolaires et au poids des origines sociales, ainsi qu'à une vision exclusive et négative de la pratique des métiers manuels. Tel n'est pas du tout le cas en Allemagne ou en Suisse, où une longue tradition est favorable à la voie professionnalisante. D'ailleurs, dans presque tous les pays de l'OCDE, à diplôme donné, les voies professionnelles permettent une meilleure insertion que les voies générales.

renforcer les savoirs fondamentaux, qui sont des utiles à tout citoyen éclairé. Il est essentiel d'accompagner cette dimension. Nous souhaitons également que le lycée professionnel soit au centre des enjeux compétences pour les filières dont la Nation aura besoin demain. Il est essentiel que les lycées professionnels puissent penser le monde économique de demain et préparer leurs élèves à ces enjeux. Ces élèves doivent

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec la massification de l'accès au baccalauréat dans les années 1980, il est apparu nécessaire d'offrir une pluralité d'orientations correspondant, dans dans la mesure du possible, à la diversité des profils des chères têtes blondes de notre pays. Avec le bac professionnel, il s'agissait de proposer une formation un peu moins théorique dans le champ de l'enseignement général et de la compléter par un enseignement professionnel de nature à encourager des vocations dans les métiers dits manuels. Chacun le sait, en réalité, il s'agit souvent d'une orientation par défaut, lorsqu'on estime que l'accès au baccalauréat général est impossible. La filière est considérablement déconsidérée par les familles et largement méconnue par les enseignants, qui sont pourtant chargés de cette orientation L'ambition était belle, mais, quarante ans plus tard, le constat est amer pour Daniel Bloch, « père » du bac pro en 1985, que je cite : « baisse significative du niveau des élèves entrant dans l'enseignement professionnel »,

Il y a la vision jupitérienne, celle qui consiste à dire à l'avance et précisément ce qu'il convient de faire, tout en convoquant une énième forme de concertation, chargée bien sûr de valider ces propositions. Qui peut raisonnablement s'étonner des réactions négatives qui escortent ce mode de fonctionnement politique, cette forme de management par imposition d'une vérité divine ? Il y a la vision arithmétique, qui consiste à traduire le nombre d'heures d'enseignement général supprimées par son équivalent en nombre de postes de fonctionnaires, 7 000 à 8 000 selon Daniel Bloch, nombre lui-même converti en économies budgétaires réalisées sur une année ou un quinquennat. Je ne veux pas croire qu'une telle démarche puisse guider à elle seule une réforme de notre système éducatif Il y a la vision syndicale, celle qui considère que tout projet de réforme porte atteinte aux statuts de la corporation et qu'il convient donc de s'y opposer fermement, parfois avant même d'être sollicité. Quelques syndicats ont néanmoins accepté de participer aux discussions et aux premiers ateliers de travail, tout en soutenant les mobilisations du 18 octobre dernier et du 17 novembre prochain.

Il y a la vision économique, qui consiste à identifier chaque élève de la filière professionnelle comme un potentiel futur candidat à l'embauche dans le secteur correspondant à sa formation. Les entreprises n'ont certes pas à définir elles-mêmes les attendus de chaque cursus, mais nous serions irresponsables si nous fermions les yeux sur le financement massif de certaines impasses, notamment dans le secteur tertiaire. Identifier les besoins ne signifie pas les traduire sur la carte scolaire, mais il s'agit bien d'un paramètre important. Il y a enfin la vision territoriale, celle des régions, qui apparaissent, me